Quand l’enfance est brisée, quand l’innocence et la confiance sont trahies, le temps n’efface rien. Il ne répare pas. Il condamne seulement à survivre, à porter des blessures invisibles, parfois sans voix, et trop souvent sans justice. Les agresseurs savent ce qu’ils font : ils élaborent des stratégies redoutables pour enfermer leurs victimes dans le silence et dans l’oubli, et les y emmurer durablement. La première de ces stratégies est au cœur même de l’inceste. En s’attaquant à nos enfants, vulnérables par nature, les agresseurs le savent : ils ciblent des victimes pour lesquelles il est impossible de parler. Parce que les agresseurs sont ceux en qui l’enfant devrait avoir le plus confiance : parents, grands parents, frères, oncles, amis de la famille, figures d’autorité. Parce qu’ils fabriquent une fausse normalité, isolent leur proie, la dévalorisent, inversent la culpabilité et verrouillent la parole. Pris au piège, l’enfant est prisonnier. Prisonnier de la sidération, qui fige son corps et son esprit. Prisonnier de la confusion, incapable de nommer l’horreur qu’il subit. Prisonnier du silence, pétrifié par la peur des représailles, du rejet, de la perte d’un prétendu « lien privilégié », de la destruction de la famille. Ce silence est non un choix, mais une impossibilité, une impossibilité que les bourreaux exploitent à leur avantage. Mais si un enfant ne verbalise pas forcément, il peut quand même s’exprimer. Il envoie des signaux que nous, adultes, devons savoir décrypter : troubles du comportement, du sommeil, de l’alimentation. C’est pourquoi j’ai déposé, au nom du Gouvernement, un amendement visant à rendre obligatoire la formation à la détection des abus sexuels pour tous les professionnels au contact de nos enfants : enseignants, soignants, éducateurs, travailleurs sociaux, animateurs culturels et sportifs, qui doivent devenir autant de tiers de confiance. Nous devons systématiquement leur donner les clés pour apprendre à voir, à entendre, à détecter, à comprendre, et ce le plus tôt possible. Mais l’enfermement ne s’arrête pas là : lorsque l’enfant devenu adulte trouve le courage de parler, il se heurte à un nouveau mur. Il a fallu des années, parfois des décennies, pour se souvenir, comprendre, nommer, affronter, et au bout de ce chemin difficile, la justice lui répond « prescription ! », ce mot pudique pour dire : « Non, c’est trop tard. Les agresseurs se servent de la prescription comme d’une arme, un rempart contre toute responsabilité. Ils savent que le temps joue en leur faveur : les preuves disparaissent, les souvenirs s’estompent, la parole des victimes est contestée. Trop souvent, quand, enfin, elles trouvent la force de parler, celles ci entendent qu’elles auraient dû le faire plus tôt. Comme si c’était une simple question de volonté. Comme si elles n’avaient pas déjà été condamnées, enfermées dans la honte, la peur ou le silence. C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à tous les amendements visant à rétablir l’article 1 de la proposition de loi dans sa rédaction initiale, afin d’introduire l’imprescriptibilité en matière civile des viols commis sur des mineurs pour leur permettre, enfin, d’espérer obtenir réparation. Parce que, si l’affaire est classée sans suite pour les auteurs, elle ne l’est jamais pour les victimes. Parce que, devant un tribunal civil, les victimes pourraient démontrer les traumatismes subis et les conséquences continues de ces derniers sur leur vie professionnelle, intime, familiale, sur leur santé mentale et sur leur santé physique.

Par ailleurs, je souhaite que nous engagions une réflexion pour accélérer le circuit de réparation. En effet, aujourd’hui, l’indemnisation des victimes prend beaucoup trop de temps. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, toutes les personnes concernées ne saisiront pas la justice, mais cette possibilité, qui leur sera désormais ouverte, pourra les aider à maîtriser leur destin, ce dont elles ont profondément besoin, car les bourreaux leur ont tout imposé. Demander et obtenir justice et réparation, c’est reprendre le contrôle sur sa propre vie. Je sais les doutes qui traversent cet hémicycle, mais je vous demande de considérer ce qu’un refus, aujourd’hui, voudrait dire pour toutes les victimes, pour celles qui n’ont pas pu parler, pour celles qui attendent et espèrent que la loi change. Dans le même temps, nous devons ouvrir les yeux sur la réalité des violences faites aux femmes, qui ne se résument pas à des coups. D’ailleurs, les violences conjugales, ça ne commence jamais par des coups. Les femmes ne sont pas stupides : si on levait la main sur elles dès le premier jour, elles partiraient en courant. Non, la mécanique est plus insidieuse. Elle est méthodique, et elle est implacable. Le contrôle coercitif est une stratégie d’anéantissement. C’est un poison qui s’infiltre lentement dans l’existence, presque imperceptiblement. Il commence par une domination qui revêt les habits de l’amour, une attention qui se mue en surveillance, un intérêt qui devient flicage. Il » surveille vos allées et venues, « il » exige des comptes sur vos horaires, « il » inonde votre téléphone de messages, « il » multiplie les appels sur votre lieu de travail. « Il » trie vos relations, il les filtre, il les efface. « Il » décide avec qui vous pouvez parler, où vous pouvez aller, ce que vous pouvez porter. Il » vous isole, vous coupe du monde, de votre famille, de vos amis, de tous ceux qui pourraient être un refuge. « Il » contrôle vos finances, il vous rend dépendante. Alors, vous commencez à douter, à vous excuser, à adapter votre comportement, pour ne pas déplaire, à vous effacer. Vous regardez par dessus votre épaule, vous vérifiez l’heure, vous pesez chaque mot. Et au bout du chemin, il ne reste plus que lui. Lui seul pour « aimer », lui seul pour « comprendre », lui seul pour « protéger ». Le piège s’est refermé. C’est alors que la violence physique ou sexuelle trouve tout l’espace pour se déployer, sans résistance possible, sans témoin, sans issue. Et que l’on ne s’y trompe pas : le contrôle coercitif ne connaît ni statut ni milieu social. La France ne peut plus ignorer cette mécanique implacable, cette stratégie qui broie les femmes et laisse les bourreaux impunis. Nous avons le pouvoir d’agir, donc nous avons le devoir d’agir. Je salue la manière avec laquelle la commission des lois a travaillé sur l’article relatif au sujet que je viens de mentionner, et je suis favorable Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, il a trop longtemps été exigé des victimes qu’elles se battent seules, trop longtemps été attendu qu’elles trouvent la force de dénoncer, d’affronter, de survivre. La lutte contre les violences ne peut plus être leur fardeau à elles. Elle doit être notre responsabilité. La République doit entendre toutes les victimes, déjouer toutes les stratégies des agresseurs et les sanctionner implacablement. Tel est notre combat, et aujourd’hui, ensemble, nous pouvons gagner une nouvelle bataille. La parole

mes chers collègues, l’intervention du législateur en matière de violences sexuelles, sexistes (VSS) et intrafamiliales est abondante. Il faut s’en réjouir, parce qu’elle est utile, nécessaire, même, et souvent saluée. Cependant, il reste encore beaucoup à faire, car le droit peine à saisir la particularité de ces infractions de l’intime. la justice rencontre de grandes difficultés à caractériser des faits qui se déroulent le plus souvent à huis clos, à l’abri des regards. Nous avons donc, Elsa Schalck et moi même, accueilli favorablement la proposition de loi déposée par Aurore Bergé lorsqu’elle était députée. Dans le bref délai qui nous est imparti, nous nous concentrerons sur deux aspects du texte : les modifications envisagées au régime de la prescription de certaines infractions sexuelles, que j’aborderai, puis la prise en compte législative du phénomène de contrôle coercitif, qu’Elsa Schalck évoquera. L’article 1 visait à introduire l’imprescriptibilité civile, et non pénale – j’y insiste –, pour les violences ou agressions sexuelles commises sur des mineurs. Comme vous le savez, seule l’imprescriptibilité pénale est prévue en droit français, et uniquement pour le génocide et les crimes contre l’humanité, même si l’action civile peut être engagée devant le juge pénal à cette occasion. L’imprescriptibilité est donc, par nature, exceptionnelle, grave, voire solennelle. L’article 1 a été supprimé par l’Assemblée nationale en commission, et n’a pas été rétabli en séance. Si la commission des lois du Sénat a maintenu cette suppression, des amendements ont été déposés pour le rétablir. Cette question, délicate politiquement et complexe juridiquement, justifie donc quelques développements avant leur examen. Je tiens à préciser que nous partageons les constats de ceux qui appellent à l’allongement du délai de prescription, voire à l’imprescriptibilité. En effet, les victimes ont souvent besoin de plusieurs années, parfois de décennies, pour dénoncer ce qu’elles ont subi et même, pour certaines d’entre elles, pour le réaliser. De plus, elles éprouvent souvent le besoin, pour se reconstruire, d’obtenir du juge la reconnaissance du dommage qu’elles ont subi. Néanmoins, nos nombreuses auditions nous ont convaincues qu’une modification trop large des règles de prescription entraînerait plus de difficultés qu’elle n’en résoudrait, et qu’elle se ferait au détriment des victimes. Ce constat est tout d’abord fondé sur la nature de la preuve, en matières civile comme pénale. La disparition des preuves dans le temps rendrait l’imprescriptibilité souvent théorique, donc déceptive, pour les victimes : nous les exposerions alors à un espoir immédiatement démenti par les faits, car elles n’auraient à apporter à l’audience que des souvenirs, sans aucune preuve matérielle. La deuxième raison découle des particularités de l’action en responsabilité civile. Je tiens à insister sur ce point, d’apparence technique, mais qui est essentiel. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, l’action en responsabilité civile se distingue par certaines spécificités qui ne sont pas favorables aux victimes, notamment parce que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Ce dernier, donc la victime, doit ainsi prouver non seulement la réalité des faits qui ont causé son préjudice, mais aussi l’existence d’un lien direct entre le dommage subi et le préjudice qui en découle. En d’autres termes, les victimes devront démontrer que leur traumatisme découle directement et uniquement des violences sexuelles qu’elles ont subies. Accepter cette situation, c’est exposer les victimes au risque de voir leur vie privée déballée, au cours de l’audience, par la défense, puisque celle ci voudra démontrer que les violences vécues, à supposer qu’elles soient établies, ne sont pas la cause unique de la souffrance psychique ressentie. C’est donc créer le risque d’un nouveau traumatisme, sans aucune garantie de réparation. Mes chers collègues, il y a là une question de principe. Voulons nous nous contenter de symboles, même si nous savons que leurs répercussions sont douteuses ? Voulons nous passer un message aux victimes, alors que nous savons qu’il sera sans portée concrète ? Un autre élément mérite d’être souligné. Contrairement à l’action publique, l’action civile en réparation se transmet aux héritiers de la victime, même si elle n’a pas été engagée avant le décès de cette dernière. Tout allongement du délai de prescription civile et,, l’imprescriptibilité, présenterait donc un risque considérable pour la paix sociale. Plus encore, il me semble que ce procédé s’apparenterait à une poursuite indéfinie, y compris par des tiers, d’une forme de réparation susceptible de s’éloigner dangereusement de l’infraction initiale. La limite entre la justice et la vengeance s’en trouverait brouillée, en même temps que les principes fondateurs de notre droit de la prescription. Voilà pourquoi la commission des lois a préféré, en matière civile, ne pas modifier le droit en vigueur. Le même raisonnement a présidé à nos choix sur l’article 2 de la proposition de loi, qui apportait plusieurs modifications aux articles relatifs au mécanisme de la prescription glissante au sein du code de procédure pénale. Si la commission est favorable à l’objectif visé par le mécanisme de la prescription glissante, qui permet de mieux appréhender les criminels en série et de réparer les préjudices du plus grand nombre possible de victimes, elle a toutefois fait preuve de vigilance pour plusieurs raisons.

chers collègues, le texte transmis au Sénat comportait des difficultés certaines. La rédaction adoptée par les députés, fondée sur les sentiments de la victime et mobilisant des termes inconnus de notre droit, présentait un risque

Pis encore, une telle création aurait produit un effet d’éviction pour les infractions existantes, y compris pour des délits assortis d’une peine plus élevée que celle qui est envisagée pour le contrôle coercitif.

Notre devoir est de prendre en considération les besoins des praticiens, qui doivent pouvoir qualifier le contrôle coercitif au cas par cas, avec une latitude qui n’exclut pas la rigueur, mais qui permet de protéger au mieux les victimes. Je tiens à insister sur une idée importante : le mieux est parfois l’ennemi du bien. À trop vouloir préciser la loi, on obtient souvent l’effet inverse à celui que l’on recherche. Entrer dans les détails ne permet pas forcément de mieux protéger la société.

Il me reste quelques instants pour évoquer un autre sujet essentiel : celui des circonstances aggravantes en matière de viol. Cet enjeu n’a pas fait l’objet de débats publics aussi nourris que l’imprescriptibilité ou le contrôle coercitif.

aux victimes de ne plus hésiter à porter plainte. En effet, nous ne devons pas oublier que le principal obstacle à la répression des violences sexistes et sexuelles tient davantage à la société elle même qu’à la loi. Le chemin est encore long pour que la honte change de camp, mais nous devons, toutes et tous, contribuer à accélérer la marche. Mes chers collègues, c’est ce que nous ferons aujourd’hui en comblant les lacunes de notre droit, sans renoncer aux principes supérieurs qui doivent guider notre action de législateur. La parole

Publié en novembre 2023, le rapport de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants présentait des chiffres absolument alarmants. 14,5 % des femmes et 6,4 % des hommes de 18 à 75 ans auraient ainsi été confrontés à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, soit 5,4 millions de personnes.

90 % des victimes développent des troubles de stress post traumatique. Or, malgré la gravité de ces violences et leurs effets sur le long terme, leur dénonciation est particulièrement difficile. Plus l’agresseur est proche de la victime, ce qui arrive souvent dans le cas des violences sexuelles contre les mineurs, plus cette dernière peine à dénoncer son bourreau. Ainsi, lorsque l’auteur des faits est un

allongé de vingt à trente ans le délai de prescription en matière pénale des crimes sexuels commis sur les mineurs. En matière civile, en l’état actuel du droit, le délai de prescription

où, en raison du délai écoulé entre les faits et le procès, les preuves sont nécessairement plus complexes à réunir. C’est pourquoi l’imprescriptibilité en matière civile, à plus forte raison quand la victime est mineure, prend tout son sens. Elle permet à la victime d’obtenir justice, la reconnaissance du préjudice subi. L’article 2 de la proposition de loi permet également à la victime de disposer de davantage de temps pour poursuivre son bourreau, grâce au mécanisme de la prescription glissante. La loi du 21 avril 2021 visant à mieux protéger les mineurs des crimes sexuels et de l’inceste ouvrait cette possibilité pour les victimes mineures lors des faits. Le présent texte l’ouvre aux victimes majeures. Là encore, cette mesure paraît nécessaire. Dès lors qu’une personne récidive et commet un autre viol, elle doit pouvoir être poursuivie pour tous les viols qu’elle a commis par le passé. Les délais de prescription ne doivent pas être un frein. Un autre aspect clé de ce texte est la question du contrôle coercitif. Cette notion a été théorisée en 2007 par le sociologue Evan sociologue Evan Stark. Elle a été utilisée dans cinq arrêts de la cour d’appel de Poitiers le 31 janvier 2024. Au premier abord, l’intégration de cette notion dans notre droit paraît être une bonne chose. Néanmoins, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale soulevait des difficultés juridiques, que Mme la rapporteure a rappelées. Le choix de définir une infraction autonome complexifie son articulation avec les délits et crimes déjà existants qui lui sont proches. Par ailleurs, les termes utilisés par l’Assemblée nationale pour définir le contrôle coercitif peuvent perturber son application concrète.

la répression des violences sexuelles est un enjeu complexe. Elle nécessite une mobilisation collective et des mesures efficaces. À nous, législateurs, d’agir pour aider les victimes, qui subissent des décennies durant les stigmates des infractions sexuelles commises à leur encontre. Le groupe Les Indépendants soutient donc bien évidemment ce texte. La

Une autre statistique est glaçante : toutes les trois minutes, un enfant est victime d’inceste, de viol ou d’agression sexuelle dans notre pays. Sous l’effet d’une libération salutaire notre société s’est emparée ces dernières années de la question des violences sexuelles, conjugales et intrafamiliales comme jamais auparavant. Au gré de prises de conscience aussi brutales que nécessaires, notre droit évolue pour rendre plus effective la protection des victimes de violences sexuelles et mieux réprimer leurs auteurs. Le Sénat est préoccupé depuis longtemps par ce sujet. d’une proposition de loi de Valérie Létard a permis l’instauration d’une aide universelle d’urgence pour les femmes victimes de violences conjugales.

que 42 400 personnes ont bénéficié de ce pack nouveau départ permettant de quitter le domicile de vie commune. C’est encore trop peu par rapport aux 230 000 victimes de violences conjugales : il faut faire connaître ce dispositif mieux et partout.

aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Chacun mesure la nécessité d’adapter notre droit à la réalité des traumatismes, qui, dans bien des cas, empêchent les victimes de parler avant plusieurs décennies.

L’Assemblée nationale avait supprimé l’article 1 de la présente proposition de loi, et notre commission des lois a maintenu cette suppression. Ledit article prévoyait l’imprescriptibilité civile pour les viols commis sur des mineurs.

énonce les raisons pour lesquelles cette mesure risquerait de ne servir ni les victimes ni notre système juridique. D’abord, la disparition des preuves avec le temps rendrait cette imprescriptibilité inefficace. ci serait source de désillusion pour les victimes, sur lesquelles pèse la charge de la preuve. L’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2022 fixant la consolidation du préjudice comme point de départ du délai de prescription assure une prise en compte élargie des traumatismes subis. sujet –, l’imprescriptibilité risquerait d’ouvrir la porte à des contentieux inextricables et interminables entre les demandeurs et leurs héritiers. Mes chers

En ce qui concerne la prescription pénale, notre droit a évolué de manière significative ces vingt dernières années. Les dernières réformes ont porté à trente ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs.

La présente proposition de loi étend aux victimes de viol, lorsqu’elles sont majeures, le mécanisme de la prescription glissante existant sur le plan pénal. Il s’agit d’une réponse pragmatique et adaptée, qui permettra à la justice de ne pas laisser impunis des crimes sexuels sériels. Je souhaite également dire un mot sur la notion de contrôle coercitif, au cœur de la proposition de loi. D’origine anglo saxonne, ce concept résulte en France d’une construction jurisprudentielle. À l’instar des arrêts de la cour d’appel de Poitiers du 31 janvier 2024, plusieurs juridictions le définissent comme « une atteinte aux droits humains en ce qu’il empêche […] de jouir de ses droits fondamentaux comme la liberté d’aller et venir, de s’exprimer, de penser, d’entretenir des liens familiaux

dans notre ordonnancement juridique. La commission des lois du Sénat a invoqué le risque constitutionnel sous jacent au concept de « contrôle coercitif » en tant qu’infraction pénale autonome. Le choix a été fait de prendre appui sur le code pénal, notamment sur l’infraction de harcèlement moral du conjoint. Dans l’intérêt des victimes, je pense que ce choix est judicieux, car il apporte une plus grande sécurité juridique. Au delà de sa qualification, le repérage du contrôle coercitif est un enjeu clé, car ces violences du quotidien, souvent invisibles, isolent progressivement les victimes. Les détecter est d’autant plus difficile que l’emprise pousse ces dernières à minimiser leur souffrance. Les travailleurs sociaux, les personnels de l’éducation nationale et les professionnels de santé doivent être formés à identifier ces signaux. Leur rôle est essentiel pour briser l’isolement. Nos débats s’annoncent particulièrement riches. Comme toujours, notre boussole doit être l’efficacité concrète des mesures que nous adopterons pour mieux protéger les victimes et mieux réprimer les auteurs de ces agressions inqualifiables, dans la rigueur

Huit ans après le début du mouvement MeToo, il y a certes eu des progrès notables, une prise de conscience collective et des évolutions législatives, mais le chemin reste encore long. La loi du 3 août 2018 est venue réprimer les violences sexistes et sexuelles du quotidien, comme les sifflements dans la rue, les remarques sexistes ou les propositions sexuelles. Cette loi a aussi porté le délai de prescription concernant l’infraction de viol sur mineur à trente ans, contre vingt ans auparavant. La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a créé de nouvelles infractions sexuelles. Aucun adulte ne peut désormais se prévaloir du consentement sexuel d’un mineur de moins de 15 ans, ou de moins de 18 ans en cas d’inceste.

C’est aussi la preuve que les magistrats se sont pleinement saisis des outils que la loi leur offre pour mieux sanctionner les auteurs. C’est aussi le signe que notre système est perfectible. Le combat contre les violences conjugales et sexuelles rencontre encore des obstacles que la présente proposition de loi a pour objet de surmonter. Tout d’abord, les règles de prescription dans le droit actuel peuvent faire obstacle à une lutte efficace contre ces violences. Il existe en effet un écart substantiel entre le nombre de victimes de violences sexuelles et le nombre de condamnations. condamnations. Dans certains cas de violences sexuelles sur mineures, la notion d’amnésie traumatique est avancée. Parfois, lorsqu’une victime trouve le courage de briser le silence, la justice lui oppose le couperet du délai de prescription, lui déniant ainsi son statut de victime au prétexte qu’elle n’a pas parlé à temps. Pour ces raisons, nous soutenons donc le rétablissement de l’article 1, prévoyant l’imprescriptibilité de l’action civile visant la réparation de violences sexuelles commises sur mineurs. Très bien ! Dans le même sens, l’article 2 de la proposition de loi instaure une prescription glissante sur les crimes sexuels commis sur les majeurs, à l’instar de celle qui est prévue pour les mineurs depuis la loi de 2021. Cette mesure permet d’empêcher que la prescription protège des auteurs récidivistes ou multirécidivistes.

pour réprimer l’accumulation d’actes qui s’inscriraient dans une stratégie de contrôle dans un couple. Pour sa part, le droit français ne comprend pas de notion équivalente. À la suite d’une jurisprudence de 2024, la proposition de loi tend à inscrire dans le code pénal une définition du contrôle coercitif. Nous soutenons cette disposition, modifiée par la commission des lois du Sénat. Un autre enjeu crucial est celui de la lutte contre la récidive des condamnés. Si tel n’est pas l’objet de cette proposition de loi, je tenais vivement, néanmoins, à en rappeler l’importance. Je souhaite que nous menions ces deux combats de front. Malgré quelques désaccords avec les positions de la commission, nous voterons naturellement en faveur de ce texte. Pour conclure, mes chers collègues, permettez moi d’avoir une attention particulière pour nos outre mer, où en 2024

il y a quelques mois, alors que je me précipite vers le métro, j’entends une femme parler au téléphone. Elle ralentit devant moi, et sa voix monte dans les aigus, marquée par une angoisse manifeste qui m’alerte. Elle parlait vite et répétait : « Je ne comprends pas ce que tu attends de moi. » Pour finir par lâcher : « Cela fait vingt quatre ans que je te préviens quand je sors du travail. Je t’appelle tous les soirs pour te dire que je rentre. Je rentre toujours directement. Je n’ai jamais été en retard. Je ne comprends pas ce que tu attends de moi. » Elle était désemparée, à bout. Sa voix, son angoisse m’ont marquée.

Le contrôle coercitif, c’est un crime contre la liberté. C’est vouloir contrôler l’autre, c’est abandonner petit à petit son autonomie, pour se rassurer, parce qu’on croit que c’est cela l’amour, pour acheter la paix, ou parce qu’on a peur.

Madame la ministre, il y a quelques jours, j’entendais une femme vous remercier de votre courage. Je m’associe à ce juste hommage. J’y ajouterai un mot : celui de pugnacité, que chacune et chacun vous reconnaît dans cet hémicycle,

il faut une expertise solide, un sol adéquat, une analyse rigoureuse, un travail d’équipe, une vision globale et à long terme, ainsi que des financements.

L’édifice pénal et civil auquel nous ajoutons quelques pierres aujourd’hui est une construction lente, parfois anarchique. Il mériterait sans aucun doute d’être remis à plat pour affirmer une politique publique claire et permettre une réponse judiciaire cohérente, lisible et, dès lors, facilement applicable par l’ensemble des acteurs. C’est pourquoi j’appartiens à la coalition parlementaire militant en faveur d’une loi globale contre les violences sexistes et sexuelles commises contre les femmes, les enfants et toutes les minorités de genre. Dans le contexte international actuel, la France s’honore en choisissant le camp de la liberté, de l’intelligence, du progrès. Vous avez réuni, madame la ministre, les représentants de tous les groupes parlementaires pour aboutir à un consensus, afin d’élaborer une réponse globale de façon transpartisane ; je vous en remercie. Il est néanmoins indispensable, une fois ce principe affirmé, de concevoir des dispositifs applicables par l’ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire, des victimes aux magistrats en passant par les forces de l’ordre, les avocats

qui, après avoir tiré dans les jambes de son ex compagne, mère de ses enfants, l’a brûlée vive. Devant de pareilles atrocités, on a envie, on a même besoin, en tant que société, de répondre de la façon la plus ferme qui soit.

Prendre en compte ces questions, c’est combattre le système qui permet la perpétuation du des violences dont sont victimes des milliers de personnes en France. Le dépôt d’un grand nombre d’amendements visant à instaurer l’imprescriptibilité civile en matière de violences sexuelles, qui n’a pas été adoptée par les députés et que nos rapporteures n’ont pas souhaité rétablir, nous permettra de débattre

essentielle, celle de prescription glissante, qui existe déjà pour les mineurs et qui sera étendue aux majeurs victimes de viol. Cette avancée considérable doit être saluée : elle permettra de juger les violeurs pour l’ensemble de leur « œuvre souvent dans des films un argument convaincre une victime de viol de porter plainte : éviter que d’autres connaissent le même sort. Cette unité sera traduite dans le code pénal et c’est une belle avancée. Il n’y a pas de solution simple. Il ne suffit pas d’adopter une mesure pour que les victimes et les acteurs judiciaires et associatifs s’en emparent ; on l’a vu avec l’ordonnance de protection. Encore faut il en effet que la mesure soit opérationnelle, lisible, constitutionnelle. Vous n’ignorez pas, mes chers collègues, que les avancées obtenues par les femmes ont comme corollaire une montée du masculinisme. J’entends moi même régulièrement des remarques agacées telles que : « C’est bon, vous l’avez obtenue, Je suis très attentive à ce mouvement de balancier, qui a toujours été observé en matière de droits humains, en particulier de droits des femmes : la réaction suit le progrès, qui reprend son cours par la suite, pour être encore de nouveau contrarié. Nous avons accompli bien des choses

Ensemble, aujourd’hui, nous décidons de porter une voix claire contre les violences sexuelles et sexistes. C’est pourquoi je suis convaincue par la nécessité d’avancer sur un sol juridique solide, qui ne puisse pas être facilement remis en cause. Mes chers collègues, le groupe Union Centriste ne fera pas défaut dans cette lutte. La parole

En 2023, les forces de sécurité ont dénombré 114 135 victimes de violences sexuelles ; 85 % des victimes sont de sexe féminin et 57 % d’entre elles sont mineures. 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France ; ainsi, toutes les trois minutes, un enfant est victime d’un viol ou d’une agression sexuelle. Nous savons cependant que ces chiffres sont largement sous estimés, puisque seulement 6 % des victimes de violences sexuelles et 14 % des victimes de violences conjugales se tournent vers les forces de sécurité.

Nous espérons que ce texte contribuera à ce que justice soit rendue et que les victimes n’aient plus à se contenter d’un classement sans suite. Je regrette néanmoins que le texte ait progressivement perdu de son ambition, notamment sur l’imprescriptibilité civile des viols commis sur des mineurs. L’enquête de la Ciivise a révélé que les faits sont prescrits pour 75 % des victimes ayant témoigné. L’abolition des délais de prescription est justement la demande la plus formulée par les victimes. Nous savons bien que de nombreuses victimes de violences sexuelles dans l’enfance n’ont pas pu porter plainte. Les raisons sont variées – menaces ou manipulations de la part des agresseurs, manque de crédit accordé à la parole des enfants ou amnésie post traumatique, phénomène bien courant

affectent durablement et lourdement la situation financière des intéressés. La prescription glissante a été instaurée en 2021 pour les viols sur mineurs. Elle permet de prolonger le délai de prescription d’un délit ou d’un crime sexuel si la même personne viole ou agresse sexuellement un autre enfant par la suite ; elle permet donc de juger l’ensemble des faits commis par des agresseurs sériels. Cela représente une avancée. Aujourd’hui, nous défendons l’extension de la prescription glissante à toutes les victimes, mineures et majeures. Nous savons que les violences conjugales ont souvent pour contexte des relations complexes, marquées le plus souvent par le pouvoir et la domination. La stratégie mise en place par l’agresseur place la victime dans une situation d’emprise, où elle se trouve privée de sa liberté et de sa capacité d’action et de défense.

Si cette proposition de loi nous met sur le bon chemin, nous resterons attentifs à la présentation d’un futur projet de loi cadre. Face au fléau des violences sexistes et sexuelles, nous devons avoir une approche globale. Les victimes doivent bénéficier d’une protection et d’une prise en charge complètes. Les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice doivent être formés, notamment à la détection des violences. Nous devons aussi augmenter les moyens de la justice civile et recruter des magistrats spécialisés dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors que nous assistons à une explosion des discours masculinistes partout dans le monde – j’espère que nous n’en entendrons pas cet après midi

Le juge Édouard Durand le rappelait : une scène de violence sexuelle n’est pas un face à face privé entre une victime et un agresseur ; elle implique un troisième protagoniste, à savoir la société, avec ses institutions. Pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, nos institutions doivent donc prendre leurs responsabilités et adopter les mesures les plus ambitieuses et les plus protectrices

les violences sexistes et sexuelles, dans les différentes formes qu’elles revêtent, sont sans doute les crimes et les délits les moins bien punis dans le monde, y compris dans les pays qui, comme le nôtre, ont choisi de les interdire En France, une femme est victime de viol ou de tentative de viol toutes les deux minutes trente, un enfant est victime de viol ou d’agression sexuelle toutes les trois minutes et trois enfants par classe sont victimes de violences sexuelles. Cette année,

Imaginons un instant que le groupe visé spécifiquement par ces violences soit un autre groupe que les femmes. Imaginons par exemple que, en France, 742 médecins

il de jours pour que les services de l’État déclarent le branle bas de combat pour mettre fin tout de suite à ce carnage ? Jamais on n’accepterait, et à juste raison, que des patients tuent un médecin tous les trois jours et qu’ils en frappent 742 par jour ! Mais, quand ce sont des femmes

Dans quelle société vivrions nous si 99,4 % des meurtres étaient impunis ? Ce constat ne constitue pas la seule particularité des violences sexistes et sexuelles.

elles sont commises par nos pères, nos oncles, nos grands pères, nos frères, nos amis, nos voisins, nos conjoints et, bien souvent, sous le regard de tous les autres. Cette spécificité des violences sexistes et sexuelles – le fait d’être victime

du point de vue de la gravité des faits commis par l’agresseur et non du point de vue de la capacité de leurs victimes à agir en justice, représentent parfois une torture qui s’ajoute au trauma.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous allons débattre aujourd’hui d’un texte attendu, qui s’attaque à une réalité que nous ne pouvons plus ignorer, mais que notre droit peine encore à saisir dans toute sa brutalité : les violences sexuelles sexuelles et sexistes. Derrière les chiffres, il y a des vies abîmées, des victimes isolées et une législation encore incapable de répondre correctement à l’ampleur de ce fléau protéiforme. La proposition de loi que nous examinons cet après midi reflète une volonté politique que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain partage pleinement. Il faut améliorer encore la protection des victimes face aux agressions sexuelles et aux violences conjugales, et durcir les sanctions prononcées plusieurs textes récents, on a progressivement renforcé la réponse judiciaire à ces violences et nous y avons pris notre part ; je pense notamment à ma collègue Laurence Rossignol, qui interviendra tout à l’heure. Au travers de ce texte, adopté par l’Assemblée nationale en janvier dernier et par la commission des lois la semaine dernière, il nous est proposé de modifier de nouveau le code pénal, le code de procédure pénale et le code civil. Nous adhérons à ces objectifs essentiels, car les violences sexuelles et sexistes continuent, évoluent et prennent des formes que notre arsenal policier et juridique doit mieux intégrer.

Oui, cela passe par une réflexion sur les délais et règles de prescription, car la parole des victimes met du temps à se libérer, non seulement quand elles ont été attaquées durant leur minorité, mais également après leur majorité. Si nous doutons de la pertinence opérationnelle et juridique de l’imprescriptibilité civile totale

J’en viens au cœur du texte, à savoir le souhait que le contrôle coercitif, un concept bien appréhendé en sociologie et « dans la vraie vie », si j’ose dire, puisse être bien appréhendé en droit ; il il est indispensable d’avancer sur ce point pour mieux protéger les victimes. Cela implique de faciliter le travail de la police, de la gendarmerie et de la justice, auprès desquelles les victimes cherchent une aide quand elles subissent des violences conjugales répétées et multiples, avec une dimension qui n’est pas nécessairement ou uniquement physique, mais qui peut être également psychologique, administrative, financière, économique. Il faut avancer, mais il faut veiller à ce que cette avancée soit, dans sa rédaction, dans sa précision, dans son interprétation, opérante en droit, sous peine d’être déceptive, voire contre productive, dans la défense des victimes et pour les professionnels qui les accompagnent. concerne l’article 3, notre groupe privilégie les contours retenus par la commission des lois du Sénat, à savoir ceux d’une infraction s’inspirant de la notion sociologique de contrôle coercitif, de la jurisprudence française récente et du droit comparé,

Nous soutenons bien évidemment l’article 5, qui répond aux attentes des associations féministes et des victimes, lesquelles dénoncent des peines parfois bien légères. Laurence Rossignol, inspiratrice directe de cette modification, y reviendra, en évoquant nos propositions d’amélioration

Pour le reste, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne veut pas que soit manquée cette occasion de renforcer par la loi la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

de donner à la justice et aux forces de sécurité les moyens concrets de faire appliquer ce droit, de mieux former les professionnels à la détection des violences sexuelles et sexistes et à leur élimination, de bien soutenir les associations qui agissent auprès des victimes, bref de prendre en compte ces violences de façon intégrale, dans toutes nos politiques publiques, afin de prévenir, reconnaître, accompagner et réparer. La parole

en 2024, seulement 104 000 femmes victimes de crime et de délit à caractère sexuel ont osé déposer plainte auprès des services de police et de gendarmerie.

de lutte contre les violences faites aux femmes ont connu une forte accélération. Sur le terrain, les progrès d’accompagnement sont tangibles, avec l’augmentation du nombre d’ordonnances de protection,

Sur le plan civil, la proposition de loi prévoyait dans sa rédaction initiale l’imprescriptibilité de l’action tendant à obtenir des dommages et intérêts en cas de viol sur mineur. L’Assemblée nationale a supprimé cette disposition. La commission des lois du Sénat a pris acte de cette suppression,

à se retourner contre celles et ceux que l’on cherche justement à protéger. En effet, toute procédure de ce type pourrait susciter de faux espoirs et engendrer des désillusions,

du classement sans suite. C’est pourquoi je n’apporterai pas mon soutien aux amendements déposés en ce sens. Sur le plan pénal, la proposition de loi examinée renforce notre arsenal juridique ; je suis convaincue que ce texte, que je voterai, porte à ce titre des avancées significatives. particulier à l’intégration, dans la définition du harcèlement sur conjoint, de faits et comportements s’apparentant à un contrôle coercitif. Je m’arrête un instant sur ce point. En ma qualité de sénateur des Français établis hors de France, j’ai créé avec Priscillia Routier Trillard et ma collègue Sophie Briante Guillemont la plateforme d’assistance Save You, destinée à venir en aide aux femmes françaises vivant à l’étranger et victimes de violences conjugales. Cela nous a amenées à examiner de près les corpus législatifs des pays étrangers en la matière, afin d’orienter au mieux les ressortissantes françaises victimes de violences conjugales. Plusieurs exemples et modèles étrangers offrent des perspectives précieuses pour faire progresser notre droit. L’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse et la Belgique ont déjà intégré dans leur législation la notion de contrôle coercitif. représente une innovation majeure dans l’appréhension de la violence conjugale, en cherchant à identifier non pas un seul acte violent, mais un schéma d’abus répétés, n’impliquant pas forcément de coups et blessures. constitue en outre un changement radical dans la logique juridique, en se centrant sur le comportement de l’auteur et non sur l’incidence de ses actes sur sa victime.

été mis en place des équipes de police spécialisées et référentes pour le suivi des dossiers, des tribunaux spécialisés pour traiter des violences de genre, tant au civil qu’au pénal, qu’une protection complète et immédiate de la victime. Les chiffres sont sans appel : le nombre de féminicides a baissé de 25 % depuis 2004 et les Espagnoles sont en proportion deux fois moins nombreuses à mourir sous les coups de leur conjoint que les Françaises.

madame la ministre, vous remercier, madame la ministre, de votre créativité juridique et de votre participation à l’élaboration de la meilleure loi possible pour protéger les femmes des violences sexistes et sexuelles.

Ces chiffres ne tiennent pas compte des violences et des féminicides contre les Françaises vivant à l’étranger. Il nous faudrait également les évaluer. Ces agressions concernent aussi des enfants et des adolescents. Les effets sont dévastateurs sur la santé physique et mentale de ces derniers, car personne ne sort indemne d’une agression sexuelle. Selon la Ciivise, 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Face à l’ampleur de ces phénomènes, cette proposition de loi – je salue l’engagement de son autrice – vise à combler plusieurs lacunes juridiques. Tout d’abord, elle nous permet de débattre d’un sujet important : l’instauration de l’imprescriptibilité civile des infractions sexuelles commises sur les mineurs. De quoi s’agit il ? En matière civile, les victimes d’infractions sexuelles peuvent demander des dommages intérêts à leur agresseur. À la différence de l’action pénale, où un agresseur est condamné à une peine pour les faits qu’il a commis, il s’agit de se tourner vers la victime de façon à tenter de réparer financièrement, s’il est reconnu, le préjudice subi.

Je comprends parfaitement les arguments avancés de part et d’autre. Ils se justifient par la douleur des victimes, douleur dont certaines ne prennent conscience que très tard, qui souhaiteraient que, d’une façon ou d’une autre, la justice leur assure : « Je vous crois.

Face à l’inévitable action du temps sur la collecte des preuves, la prescription vise à éviter de donner de faux espoirs aux victimes, même si la preuve – il est vrai – est plus simple à apporter au civil. Cela étant, les règles ont récemment évolué grâce à la Cour de cassation. Dorénavant, le délai de prescription court à compter de la date de consolidation du dommage, c’est à dire du moment où le dommage ne s’aggrave plus. Or cette consolidation peut intervenir très tard, bien après les faits. Autrement dit, la nouvelle jurisprudence permet aux victimes de faire condamner leur agresseur au civil même si les faits sont prescrits au pénal, parfois des décennies après l’infraction. Cela nous semble un compromis intelligent et suffisant, même si nous restons, bien entendu, ouverts au débat.

Le « contrôle coercitif » définit diverses stratégies de contrôle et de domination subtiles et perverses qui visent à restreindre progressivement l’autonomie et la liberté de son partenaire. Plutôt que d’en faire une infraction autonome, les rapporteures ont choisi d’intégrer les faits et comportements s’apparentant Il me semble que cette voie est juridiquement la bonne. Avec cette nouvelle définition, les autorités auront la possibilité de réprimer des comportements qui, pris isolément, paraissent anodins, mais qui font partie d’un véritable système de domination et de coercition.

surtout dans une matière qui ne cesse d’évoluer et de se nourrir des changements de notre société, de la libération de la parole et de la recherche en sociologie et en droit. La loi a évolué, la jurisprudence a évolué

ci ne peut pas être le seul. Une loi cadre, englobant des mesures à la fois sur l’éducation, la prévention, la récidive ou encore l’accompagnement des victimes, nous semble tout à fait essentielle. Le groupe RDSE aimerait d’ailleurs que soit inclus dans une telle loi l’élargissement du dispositif

vingt ans après la date de consolidation du dommage. En réalité, ce délai prive de réparation de nombreuses victimes. Les traumatismes physiques et psychiques retardent souvent la prise de conscience des violences subies. L’amnésie dissociative,

à rétablir l’article 1 pour inscrire dans le code civil l’imprescriptibilité de ces crimes. Si la justice pénale punit les coupables, la justice civile doit permettre aux victimes de faire valoir leurs droits et d’obtenir réparation. Ce point est essentiel. La procédure civile est plus souple, plus rapide et moins formelle. La charge de la preuve y est allégée. Elle permet d’obtenir réparation même sans condamnation pénale ou après un classement sans suite. Surtout, elle permet aux victimes d’être reconnues en tant que telles. D’autres pays ont déjà fait ce choix : Suisse, Pays Bas, Danemark, Belgique, Canada et Royaume Uni.

l’imprescriptibilité en matière civile pour les infractions sexuelles commises sur mineur. En effet, il faut parfois plusieurs décennies pour qu’une victime se manifeste et dénonce son bourreau. Pendant ce temps, ce dernier n’est pas du tout inquiété.

années à comprendre ce qui leur est arrivé. L’amnésie post traumatique chez les victimes de violences sexuelles dans l’enfance est fréquente. À leur âge, les enfants sont vulnérables, immatures et ne peuvent pas toujours identifier ce qui leur est arrivé ni comprendre la gravité des actes subis.

l’imprescriptibilité est conforme aux conventions internationales et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans sa résolution 2330 votée le 26 juin 2020,

Au pénal, l’action publique pour les crimes de torture, de barbarie et de viol, et pour les délits d’agression sexuelle sur mineur se prescrit par trente ans, à compter de la majorité des victimes. Certaines d’entre elles peuvent donc voir leur agresseur condamné sans obtenir réparation réparation au civil. L’amnésie dissociative n’a pas pour seul effet de retarder la prise de conscience des violences subies : elle bouleverse complètement la vie des victimes. Leur monde s’effondre. Il faut parfois des années, voire des décennies, avant qu’elles ne se sentent prêtes à s’exprimer et à entamer une démarche judiciaire. Par conséquent, cet amendement vise à rétablir une forme d’équilibre. Certes, le point de départ des délais n’est pas le même au pénal, il court à partir de la majorité de la victime ; au civil, il court à partir de la consolidation du dommage –, mais il est juste et logique d’aligner les durées. Par ailleurs, cet amendement répond à une préoccupation soulevée en commission. Contrairement à l’imprescriptibilité, il permet d’éviter une situation où, au civil, les héritiers d’un agresseur décédé seraient poursuivis à sa place. Avec un délai limité à trente ans, nous écartons le risque d’un contentieux qui se transmettrait sur plusieurs générations. Je vous propose donc cet amendement de repli qui tend à allonger le délai de prescription au civil. La parole

agir contre lui. Vous envisagez ensuite d’apporter une exception majeure au droit des successions, plus particulièrement à l’article 873 du code civil. Celui ci dispose que « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession

J’ai en mémoire l’audition du juge Durand par la délégation sénatoriale aux droits des femmes, au cours de laquelle nous avons toutes et tous été très ébranlés. L’abolition des délais de prescription, y compris au civil, répond aux attentes formulées par les victimes et par les associations qui les représentent. J’entends les arguments de ceux qui souhaiteraient maintenir la suppression de cet article 1. Mais que peuvent penser les victimes qui écoutent nos débats cet après midi ?

? Oui, monsieur le président. sommes bien d’accord, il s’agit d’imprescriptibilité civile. Et, bien entendu, les débats que nous avons là ne remettent nullement en question l’engagement des uns et des autres dans la lutte contre les violences faites aux

faites aux mineurs. Dans une décision du 24 mai 2019, ajouterai je, le Conseil constitutionnel a estimé que l’extension de l’imprescriptibilité à d’autres crimes que les crimes contre l’humanité n’est pas contraire aux lois fondamentales de la République. La parole

dit, il reste un argument de taille, qui est celui de la conservation des preuves. Comme cela a justement été rappelé tout à l’heure, l’action civile prévoit la démonstration de la réalité de faits fautifs et d’un lien de causalité entre les faits fautifs et un préjudice établi. Une telle démonstration peut être compliquée à faire pour la victime…

Toutes les trois minutes ! Quel genre de société accepte cela ? En votant ces amendements, nous poserions un interdit social.

considérablement la donne. J’ai entendu les arguments : on pourra dire à la victime qu’elle pourra potentiellement et théoriquement avoir accès à un juge.

c’est l’action qui permet à une victime de déclencher une enquête pénale, portant sur des faits constitutifs d’une infraction, c’est à dire d’un trouble à l’ordre public. Dans le cadre de cette procédure, elle pourra éventuellement obtenir aussi l’indemnisation de son préjudice. donc une action civile et une action pénale, qui sont de natures sensiblement différentes. La prescription dont il est ici question, c’est la prescription que l’on appelle « extinctive », qui consiste à laisser passer un laps de temps à l’issue duquel il ne sera plus possible pour la victime d’engager une action, donc de faire reconnaître ses droits. Cela vaut, j’y insiste, pour l’action civile comme pour l’action pénale. Il est des règles, dans le droit, qui sont purement techniques et il en est d’autres qui ont un fondement. La prescription a un fondement

n’est pas la moindre des objections à l’imprescriptibilité –, les crimes contre l’humanité et les génocides ne doivent pas être oubliés. C’est même l’inverse ! D’ailleurs, nous les commémorons régulièrement.

Il faut, comme le prévoit le code civil, que la personne qui veut agir ait connu ou ait été en situation de connaître les faits qui permettent d’agir. Le fait que le point de départ soit fluctuant ne saurait donc constituer, à mon sens, un argument de droit. La consolidation est un point de départ fluctuant,

d’un dossier qui apportera des preuves. Or il est extrêmement difficile, dans les matières dont nous parlons, d’obtenir des preuves. En revanche, en cas de plainte au pénal, l’enquête se fait

si l’auteur des faits viole ou agresse sexuellement un autre enfant par la suite. Elle permet ainsi de juger l’ensemble des faits commis par des agresseurs sériels. Pour l’heure, elle ne s’applique qu’aux victimes mineures ; nous proposons de l’étendre aux victimes majeures ayant subi un crime de viol. Une telle évolution semble nécessaire dans la mesure où, le plus souvent, le violeur ne commet pas à un seul de grandes affaires judiciaires médiatisées, récentes ou non. Nous devons conférer à notre droit les moyens de mieux réprimer ces infractions sérielles. En l’état du droit,

agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle. Cette approche est plus juste, car elle repose sur une vérité que nous connaissons tous. Dans la pratique, les viols, les agressions et les atteintes sexuelles relèvent d’un même continuum d’infractions ; l’affaire Joël Le Scouarnec illustre tragiquement cette réalité.

Une victime d’un viol subi dans l’enfance peut porter plainte au pénal jusqu’à ses 48 ans. Mais ce délai reste forcément forcément insuffisant. De nombreux témoignages montrent que certaines victimes ne retrouvent la mémoire ou ne se sentent capables de dénoncer les faits que beaucoup plus tard. En 2023, 75 % des témoignages recueillis par la Ciivise concernaient des faits prescrits. Cela s’explique par le fait que 50 % des victimes d’inceste souffrent d’amnésie dissociative. Ce n’est pas aux victimes de s’adapter au droit, mais bien au droit de s’adapter à leur processus de reconstruction. Le délai de prescription de trente ans empêche ainsi de nombreuses victimes d’obtenir justice, non parce qu’elles n’ont pas voulu parler plus tôt, mais parce que leur traumatisme les a empêchées de le faire. À ce titre, dans sa recommandation 60, la Ciivise appelle à rendre imprescriptibles les violences sexuelles commises sur un mineur. La question de l’imprescriptibilité civile, dont nous avons débattu, ne fait pas consensus. Celle de l’imprescriptibilité pénale divise tout autant, voire davantage. Je vous propose donc une voie médiane. L’amendement que je vous soumets vise à doubler le délai de prescription existant au pénal. À l’échelle internationale, d’ailleurs, la tendance est à l’abolition ou à l’allongement des délais de prescription. Aujourd’hui, dix huit

62 % des victimes de viol choisissent de ne pas informer les autorités pour éviter de revivre leur traumatisme. Le parcours judiciaire peut être une épreuve. Les victimes doivent souvent raconter leur histoire à plusieurs reprises devant différents interlocuteurs. Ces répétitions sont difficiles, elles peuvent raviver leur douleur et aggraver leur détresse psychologique. Afin d’améliorer leur prise en charge, cet amendement vise à rendre possible l’enregistrement audiovisuel des auditions de victimes majeures, sous réserve de leur accord. Le code de procédure pénale prévoit déjà cette possibilité pour les mineurs. Je vous propose de l’étendre à toutes les victimes de violences sexuelles, quel que soit leur âge. L’objectif est double : protéger les victimes et renforcer la qualité des preuves.

une circonstance aggravante du harcèlement sur conjoint. Le second intérêt est de reconnaître pleinement les effets du contrôle coercitif sur l’ensemble des victimes, y compris sur les enfants, et de donner à la justice les outils nécessaires

33 2 1 du code pénal les comportements ou les propos répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la vie professionnelle des victimes. En effet, le contrôle peut aussi passer par le fait de contraindre une personne à ne pas travailler, à l’obliger à arrêter de travailler ou à quitter une formation. On lit malheureusement

cherchent fréquemment à nuire à la vie professionnelle de leurs compagnes. Cela leur permet de maintenir leurs victimes dans une situation d’emprise, de dépendance économique et matérielle. Or c’est justement grâce à l’autonomie financière permise par la vie professionnelle qu’une victime pourra facilement, ou plus facilement, s’émanciper de son conjoint violent, et trouver de l’aide. Entraver sa vie professionnelle, c’est entraver son indépendance, sa possibilité de fuir, et de se reconstruire en cas de violence. Pour mieux protéger les victimes des violences, il me semble donc opportun d’inclure l’entrave à la vie professionnelle dans l’ensemble des faits harcelants qui restreignent leur liberté. Quel est

par la Cour de cassation dans un arrêt de sa chambre sociale du 19 octobre 2011, celle ci est un concept qui ne tient pas au rapport entre deux personnes dans un couple, mais qui « comprend l’ensemble des faits dont la relation de travail constitue la cause ». Une nouvelle fois, évitons d’inclure dans notre droit des notions étrangères qui, sous couvert de protection des victimes, auront pour effet

En effet, une menace physique permet à un conjoint de maintenir sa victime dans la peur, menaçant ainsi sa liberté et sa vie personnelle. Une femme qui vit sous la menace d’être de nouveau violentée est, de ce fait, placée dans une situation de contrôle et de captivité. Le contrôle coercitif peut s’exercer au travers de ces pressions ou de ces menaces physiques. Ces pressions permettent aux conjoints de contrôler, d’asservir la victime, au même titre que des pressions ou des menaces psychologiques ou financières.

du contrôle coercitif en prenant en considération les menaces ou les pressions numériques sur les victimes. En effet, le contrôle coercitif s’exerce également par les détournements de technologies pour organiser ou intensifier le contrôle, au travers d’une surveillance numérique avec des GPS, des logiciels espions, mais aussi du cyberharcèlement, de la manipulation d’objets connectés, de la création de fausses identités ou réalités, et de la diffusion non consentie d’informations privées. Le but est de renforcer l’isolement et la peur des victimes. Mais les agresseurs détournent aussi les outils à des fins de chantage ou de manipulation psychologique,

révèle que 42 % des femmes victimes de violences conjugales restreignent leur activité numérique pour échapper à la surveillance, ce qui a des conséquences sur leur travail et leur liberté d’expression. Nous vous proposons donc de renforcer la définition du contrôle coercitif afin qu’elle protège mieux les victimes face aux enjeux du numérique. J’ajoute qu’il est difficile est difficile d’apporter des preuves d’une fraude aux prestations sociales, d’un détournement d’allocations familiales ou d’un usage frauduleux des polices d’assurance, même

Par cet amendement, nous souhaitons remplacer la mention de pressions et menaces « financières » par celle de pressions et menaces « économiques », dont la définition me semble plus large. La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, dite convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, intègre la violence économique dans la définition des violences conjugales. Les pressions économiques du conjoint

comptes bancaires, par le contrôle total des ressources du couple, ou par la privation de ressources plaçant la femme en situation de demande, même pour les achats quotidiens de la famille. Ces pressions économiques peuvent également passer par la mise en danger du patrimoine familial et personnel de la femme. Nous savons que ces situations sont, hélas ! trop nombreuses. Le terme de « pressions et menaces économiques » présente un double intérêt. En premier lieu, il se rattache à une notion juridique déjà définie en droit international. En second lieu, il englobe davantage de situations pratiques, y compris les pressions financières. Remplacer le terme « financières » par le terme « économiques » permettra donc, selon nous, de mieux protéger les victimes.

aura pour objet ou pour effet de « contraindre la vie quotidienne de la victime ». La formulation que nous avons choisie permet de couvrir ces différents cas, notamment celui où la victime est empêchée d’utiliser normalement ses comptes bancaires,

dont la chambre sociale a établi, en 2017, qu’étaient constitutives de pressions les manœuvres tendant à faire croire à une salariée qu’elle obtiendrait la restitution de son animal de compagnie si elle démissionnait d’une entreprise.

En effet, la notion de pressions psychologiques est appréciée de manière large et plastique par les magistrats. Ceux ci ont par exemple considéré, dans un

est rédigé vient ajouter une charge probatoire qui n’a pas lieu d’être puisque, avec une telle précision, on pourrait débattre du lien affectif entre la victime et l’animal, ce qui serait source de complexité et rendrait la répression plus incertaine.

Avec cet amendement, nous proposons de compléter la définition du contrôle coercitif en considérant que « l’usage abusif

sont des circonstances aggravantes. De nombreux auteurs de violences utilisent, par exemple, le système judiciaire comme un levier pour prolonger leur contrôle coercitif après la séparation, souvent sous couvert de l’exercice de leurs droits parentaux. Ces stratégies incluent la multiplication des procédures judiciaires, des incidents procéduraux, ainsi que des actions visant à déstabiliser émotionnellement et financièrement les victimes. Je veux également insister sur l’aspect financier de telles pratiques. Les auteurs exploitent le système judiciaire, ils multiplient les recours pour imposer des coûts prohibitifs et contester systématiquement la crédibilité des victimes qui, elles, continuent de se mettre à nu et de raconter leur vie. Ces tactiques servent non seulement à prolonger le conflit, mais aussi à maintenir un contrôle sur les victimes, avec des répercussions sur la santé de ces dernières, leurs ressources, leur activité professionnelle et leur liberté. Cet amendement a donc pour vocation d’aggraver la sanction lorsque ces procédures sont utilisées par les auteurs du contrôle coercitif,

dans les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à l’ordonnance de protection et au consentement contractuel. Quel

de prendre en considération les comportements s’apparentant au contrôle coercitif. Le code civil mentionne explicitement les violences psychologiques parmi les éléments au regard desquels le juge se détermine. La magistrate Gwenola Joly Coz elle même, que l’on ne saurait soupçonner d’être opposée à la reconnaissance du phénomène – si nous sommes réunis aujourd’hui, en effet,

pose l’exercice de la justice aux affaires familiales dans les situations de contrôle coercitif. Nous serons confrontés à des situations dans lesquelles le contrôle coercitif, ou le harcèlement, tel qu’il est défini, ne sera ni jugé par le juge pénal

appliquées, opérationnelles, et qu’elles protègent efficacement les familles.

d’ores et déjà des circonstances aggravantes pour le crime de viol, notamment lorsque la victime présente une vulnérabilité particulière. Toutefois, cette disposition ne couvre pas spécifiquement les agressions commises dans un établissement de santé. Pourtant,

Plusieurs dépôts de plainte ont été enregistrés au cours des dernières années, et ces affaires ne sont pas isolées. Les victimes peuvent être agressées par d’autres patients, par des personnes extérieures, voire, parfois, par le personnel soignant, comme l’a tragiquement illustré l’affaire Dans les établissements de santé mentale, la vulnérabilité est extrême. Certains patients sont attachés à leur lit dans une chambre dont la porte reste ouverte ; ils sont sans défense, livrés à d’éventuels agresseurs. Dans ces conditions, la violence sexuelle prend une dimension encore plus

madame la rapporteure.

procède du constat qu’un nombre croissant de viols sont filmés par leurs auteurs, puis diffusés, notamment en ligne, sans que notre droit permette de sanctionner pleinement ces agissements. Notre

Cette hypothèse n’est prise en compte qu’au titre de la complicité ; or, comme vous le savez, on ne saurait être à la fois auteur et complice. Il s’agit là d’une lacune regrettable que nous avons aujourd’hui l’occasion de combler. Nous remercions donc Mme Billon et l’ensemble des cosignataires d’avoir déposé cet excellent amendement

favorable sur cet amendement.

à faire usage de ce mécanisme dans une situation de contrôle coercitif. Nous ne pouvons en effet ignorer que celui ci s’inscrit très fréquemment dans une escalade de violences qui peut se terminer tragiquement par un féminicide. L’urgence de telles situations justifie pleinement d’étendre ce nouveau régime de protection à ces situations alarmantes afin de protéger au mieux les victimes.

à libérer la parole, régulièrement reprise dans les campagnes de sensibilisation et de prévention sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants, peut être faudrait il

relatifs à l’ordonnance de protection, j’avais regretté que les violences économiques soient insuffisamment prises en compte dans le cadre des mesures que le juge aux affaires familiales peut